l'économie sociale et solidaire, ou ESS, regroupe l'ensemble des structures économiques dont le statut, l'organisation, le fonctionnement et l'activité sont fondés sur les principes de la solidarité, de l'équité et de l'utilité sociale. Leur objectif est de favoriser la création d'emplois dans une perspective d'insertion ou de réinsertion, ainsi que d'une plus grande cohésion sociale. Principalement constituées en associations, en mutuelles, en coopératives ou en fondations, les entreprises de l'ESS adoptent des dispositifs de gestion et de décision participatifs et démocratiques, avec un encadrement strict de l'utilisation des résultats financiers - pas de profit personnel, réinvestissement des bénéfices. Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nombre de nos concitoyens participent ou ont affaire à des entreprises de l'ESS sans s'en douter. Ce déficit de notoriété, auprès des citoyens comme des décideurs politiques, est bien l'un des soucis majeurs de ce qui peut être considéré comme un modèle économique alternatif et différent. De plus, si certaines des entreprises de l'ESS répondent à ces principes originels, d'autres, au fil du temps, ont eu tendance s'en éloigner ou,, à moins les brandir en étendard. Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas d'une sorte de reproche, car toutes les entreprises de l'ESS partagent toujours ces principes, derniers ne sont souvent ni rappelés ni connus des nouvelles générations et de nombre de décideurs, la perte de reconnaissance amenant ainsi à une perte de connaissance. Aussi, au travers de ce débat, souhaité par le groupe GEST, nous souhaitons mieux faire connaître ce que porte et représente l'ESS, alerter sur la fragilisation de ses structures pendant la crise sanitaire et sur sa place dans les plans de relance économique, et, enfin, formuler des propositions lui permettant de peser de tout son poids dans la perspective de la transition écologique, sociale et solidaire qui nous apparaît impérative. Les différents acteurs de l'ESS se sont donc structurés peu à peu pour défendre et promouvoir ses valeurs et encourager son financement par la mise en place de partenariats, tant publics que privés. En France, parmi les organisations les plus représentatives, on peut citer le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, le CNCress, le Mouvement associatif, Coop FR, qui est le mouvement des coopératives, le Mouvement des entrepreneurs sociaux, ou Mouves, la Fédération nationale de la mutualité française, et j'en Le poids économique est de plus en plus significatif : 2,4 millions de salariés, dont 68 % de femmes ; 22 millions de bénévoles ; 222 000 structures labellisées ESS ; 10,5 % de l'emploi total ; 14 % des emplois privés ; 10 % du PIB ; 35 millions d'adhérents à une mutuelle de santé. Dans les Dans les territoires fragiles, elle représente 22 000 établissements et 161 000 salariés en milieu rural, ainsi que 10 000 établissements et 104 000 salariés dans les quartiers de la politique de la ville. Le modèle le plus connu, celui de la coopérative, est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. La coopérative est un des uniques modèles économiques qui permette réellement de concilier performance économique, respect de l'humain, gouvernante démocratique, création d'emplois durables et innovation. noter le cas unique de Railcoop, une entreprise ferroviaire, et les expériences de coopératives créées par les travailleurs après une faillite ou un conflit social, comme Scop-Ti, producteur de thés à Gémenos, symbole de la pérennité des coopératives se substituant à des entreprises capitalistes classiques qui se mettent en faillite. En 2018, quelque 22 600 entreprises coopératives en France emploient 1,3 million de salariés. La loi du 31 juillet 2014 relative à l'ESS, complétée en septembre 2016, est destinée à fixer et consolider les règles et la gouvernance de l'économie sociale et Elle ouvre notamment l'ESS aux structures à statut commercial, optant pour ses principes et intégrant des objectifs d'utilité sociale. La loi prévoit en outre un dispositif d'agrément réactualisé dit « ESUS ». Elle marque la reconnaissance législative « d'un mode d'entreprendre différent Elle permet notamment de définir clairement une organisation nationale et régionale de l'ESS. Il apparaît essentiel de ne pas toucher à ce socle légal. La crise sanitaire a vu, comme pour l'ensemble des acteurs économiques, les activités et les emplois de l'ESS fortement touchés, notamment dans les secteurs des services d'action sociale, de l'éducation et des services à la personne. Le secrétariat d'État a mobilisé un fonds d'urgence de 30 millions d'euros pour les structures du secteur de moins de 10 salariés. Pour autant, plus globalement, d'après vos propres chiffres, madame la secrétaire d'État, l'ESS ne pèse que 1,3 milliard d'euros

Les Cress ont dû développer des relations avec les conseils régionaux. Cela représente l'avantage d'une meilleure adaptation territoriale, mais a pour conséquence de rendre difficile une consolidation à l'échelle nationale de leurs données, notamment dans l'analyse et la qualification des besoins des entreprises de l'ESS. Nous jugeons indispensable un renforcement des crédits déconcentrés, pour assurer le financement de ce socle et ouvrir de nouvelles actions d'accueil, d'information et d'orientation permettant de consolider la qualification de la chaîne de l'accompagnement à l'échelle nationale. Il est également nécessaire d'établir un état des lieux périodique du financement de l'ESS, qui en décrirait les caractéristiques et tendances, estimerait les besoins de financement futurs par famille et secteur, et, enfin, suggérerait les adaptations. Cet état des lieux requiert la mise à disposition par l'administration de données en. Par ailleurs, il importe de garantir l'accessibilité aux dispositifs ouverts aux entreprises commerciales pour toutes les entreprises de l'ESS. Il devient aussi urgent de rappeler aux décideurs publics que de nombreuses entreprises de ce secteur ne bénéficient pas forcément de l'agrément ESUS.

Le mouvement associatif, acteur important de l'ESS, a souligné un fort taux de non-recours aux dispositifs de soutien mis en place, en raison non seulement de l'inadaptation de certains dispositifs, mais également de difficultés d'accès à l'information et du manque d'ingénierie pour la recherche et l'obtention de ces financements.

de l'ESS, en permettant aux associations dont l'activité dépend d'une tarification publique ou de subventions pour délégation d'action la mise en réserve d'une partie de leur résultat d'exploitation. Au-delà, mieux financer l'innovation sociale doit être au coeur de notre réflexion. Nous pourrions par exemple envisager de favoriser la reprise d'entreprise, notamment dans le cas de départ à la retraite de l'employeur. Là encore, cela nécessiterait plus de moyens pour les Cress.

d'utilité sociale agréées

et le devenir de notre économie sociale et solidaire. Cela faisait plusieurs années que ce débat ne pouvait se tenir, et pour cause : il manquait un portage gouvernemental et une ou un ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

C'était d'autant plus important que la représentation de l'ESS au Gouvernement a quasiment coïncidé avec le début d'une crise sanitaire, qui s'est très vite muée en une crise économique, laquelle met encore à rude épreuve les structures de l'économie sociale et solidaire, comme le reste des entreprises conventionnelles. En effet, cette crise

S'y ajoute un accès limité aux financements bancaires et publics. L'exemple symptomatique est bien sûr celui des petites associations employeuses, qui, d'un côté, subissent la réticence des banques, et, de l'autre, ne connaissent pas forcément les dispositifs d'aides de l'État ou estiment même parfois, voire trop souvent, qu'ils ne leur sont pas destinés. C'est le premier chantier auquel j'ai souhaité m'atteler en arrivant l'été dernier à Bercy. Pour reprendre l'expression de M. le sénateur Benarroche, de M. le sénateur Benarroche, ce manque de connaissance, parfois même des acteurs publics, ce manque de reconnaissance, aussi, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, m'ont conduit à répondre d'abord et avant tout à l'urgence, en luttant contre le non-recours. Depuis juillet dernier, nous avons successivement mis en place un guide pour expliquer à l'ensemble des acteurs de l'ESS comment bénéficier des aides d'urgence, mis à jour l'ensemble des informations pour recenser tous les appels à projets du plan de relance qui concernent l'ESS, et fait en J'imagine le sourire goguenard que peut susciter l'évocation même d'un numéro vert, mais je connais aussi très bien la détresse de l'employeur qui ne trouve pas de réponses à ses questions. J'ai donc non

J'ai donc non seulement souhaité que les services de l'État disposent des réponses susceptibles d'être posées par les acteurs de l'ESS, mais aussi très directement missionné mon cabinet, pour garantir aux acteurs des réponses à leurs questions, si tant est qu'ils ne les aient pas trouvées par les autres moyens mentionnés. puis vous assurer que c'est le cas très souvent. Depuis le début de la crise, je me mobilise, avec Bruno Le Maire, pour rappeler que les structures de l'ESS sont très simplement des acteurs économiques à part entière, et que, de ce fait, tout aussi simplement, elles sont légitimes à être éligibles à toutes les mesures de droit commun. C'est le cas aujourd'hui. Je ne le sais que trop bien, les spécificités de l'ESS la rendent plus fragile, et les mesures de droit commun peuvent se révéler soit mal calibrées, soit insuffisantes, voire, je le répète, trop souvent méconnues par les structures mêmes de l'économie sociale et solidaire. C'est ce fameux non-recours contre lequel je me bats.

qui permet, dans nos territoires, de soutenir le recours des associations à des prestataires externes pour se développer et mieux répondre aux appels à projets. C'est pourquoi, enfin, j'ai fait voter en collectif budgétaire, et vous l'avez mentionné, monsieur Benarroche, le fonds UrgencESS, doté de 30 millions d'euros, à destination des petites structures employeuses de l'ESS. Avec ce fonds, nous souhaitons toucher tous les acteurs, surtout ceux qui n'ont pas coutume de demander des aides publiques ou à qui elles ont été refusées. Aussi, j'ai fait en sorte qu'il soit le plus simple d'accès possible. Il a été confié à un acteur que vous connaissez bien, et qui connaît bien les territoires, à savoir France Active. Il a un fonctionnement très simple un guichet unique sur urgence-ess.fr ; un diagnostic simple individualisé, qui permet d'identifier les aides de droit commun auxquelles la structure peut prétendre ; une subvention allant de 5 000 à 8 000 euros en fonction des besoins, ainsi qu'un accompagnement renforcé par le DLA pour les structures éligibles.

7 373 structures avaient fait une demande sur le portail ; 4 534 dossiers sont en cours d'instruction, et, aujourd'hui, ce sont 1 600 dossiers qui sont déjà en cours de traitement pour cette aide d'une première tranche de 10 millions d'euros. Ce mouvement est important de préciser que, pour les deux tiers, il s'agit d'acteurs qui n'étaient jusqu'à présent pas identifiés par France Active. Il y a ainsi des acteurs qui sollicitent des aides pour la première fois. Il y a deux manières de considérer cette réalité : c'est à la fois un sujet d'inquiétude, car cela montre la grande fragilité de notre tissu économique social et solidaire, mais c'est aussi un motif relatif de satisfaction, parce que cela veut dire que ce combat contre le non-recours que nous menons commence tout juste à porter ses fruits. Quoi qu'il en soit, j'entends poursuivre le travail pour que le « quoi qu'il en coûte » s'applique à l'économie sociale et solidaire. À mon sens,

comme l'économie circulaire, les ressourceries, les recycleries, le secteur médico-social ou le soutien à l'emploi des personnes en situation de handicap. Je crois profondément que l'ESS a un avenir, non pas juste pour elle-même, mais pour toute notre économie. mais pour toute notre économie. Ce n'est pas le débat de ce soir, certes, mais force est de constater que les pratiques de notre économie sociale et solidaire sont en train d'essaimer dans notre économie. Nous le voyons sur la gouvernance, qui se démocratise, sur la limitation des profits, sur la prise en compte de l'impact écologique et social des activités économiques. C'est cette influence que je souhaite aider l'ESS à valoriser. C'est d'ailleurs, et j'en terminerai sur ce point, la philosophie des contrats à impact que j'ai relancés au début de mon mandat. Il s'agit d'une nouvelle source de financement pour les acteurs

Certes, nous devons encore tout faire pour aider l'ESS à passer la crise. Toutefois, je partage avec vous, sincèrement, la conviction que l'économie sociale et solidaire nous aidera à nous dépasser par la suite. Nous allons au débat interactif. Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, suivie d'une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial

sociale ? La consommation durable se situe à l'intersection de ces modèles économiques. C'est sur ce point que je souhaiterais attirer votre attention, et plus particulièrement sur le reconditionnement des produits d'occasion. Dans le cadre des débats autour de la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, le Gouvernement a avancé la possibilité d'assujettir les produits d'occasion reconditionnés à la redevance « copie privée Cette taxe a été créée en 1985 pour compenser un manque à gagner des ayants droit sur les produits copiés. Si elle était appliquée, le secteur français de l'économie circulaire pourrait connaître une perte estimée à plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. S'il semble légitime de protéger la culture, cela ne doit évidemment pas mettre en péril l'emploi local ou les modes de consommation responsable. En effet, l'économie circulaire a permis la création en France de plus de 5 000 emplois, notamment dans des entreprises du secteur marchand et des organisations solidaires intégrant des personnes en formation, en insertion, en situation de handicap. En outre, le reconditionnement, c'est permettre de prolonger la durée de vie d'un produit et, partant, éviter d'utiliser davantage de matières premières afin de produire de nouveaux biens. Enfin, reconditionner, c'est rendre accessible au plus grand nombre les nouvelles technologies de l'information et de la communication, puisque plus de 70 % des Français achètent régulièrement des produits d'occasion. au regard de ces implications, à la fois économiques et environnementales, la redevance pour copie privée sur les produits d'occasion reconditionnés est-elle vraiment pertinente ? La parole est à Je vous remercie, monsieur le sénateur Gold, de souligner l'importance de la filière du reconditionnement. C'est en effet pour moi l'exemple même de ce que nous voulons faire en matière de croissance verte, c'est-à-dire une croissance fondée non seulement sur la baisse de notre empreinte carbone, mais aussi sur un emploi de proximité. Le Parlement examinera bientôt, vous le savez, le projet de loi « climat et résilience », dont plusieurs dispositions vont précisément venir encourager les acteurs de cette croissance verte, que ce soit dans l'alimentation, le bâtiment ou, bien sûr, la réparation, avec l'obligation de mise à disposition de pièces détachées. Dans ces conditions, je ne puis que vous confirmer le plein soutien du Gouvernement à ce secteur du reconditionnement. Quelques start-up françaises s'y affirment de plus en plus, et il faut, je crois, s'en féliciter, parce que cela montre

des entreprises d'insertion, qui sont d'ailleurs souvent sollicitées par ces nouvelles plateformes. L'enjeu est de taille, comme vous l'avez rappelé. L'électronique reconditionnée pourrait créer dans les années à venir plus de 20 000 emplois, sachant que, pour chaque téléphone reconditionné, c'est l'équivalent de 30 kilogrammes de CO2 évités. À l'heure actuelle, je crois que le débat est essentiellement juridique. Il s'agit en réalité de savoir si un portable reconditionné est mis sur le marché ou remis sur le marché, ce qui est le premier déterminant de la redevance « copie privée C'est la question qu'il faudra trancher et sur laquelle les réflexions, à cette heure, sont encore en cours. Mon cabinet suit évidemment cela de très près. J'ai aussi, bien évidemment, mon opinion personnelle, mais vous comprendrez aisément, au risque de finir par une pirouette, qu'en tant que secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire je me devrai d'être solidaire de la position qu'adoptera finalement le Gouvernement sur cette question, dont je maintiens

L'économie sociale et solidaire est touchée par la crise, comme bien d'autres secteurs. Mais, d'une certaine façon, elle constitue une voie de sortie de cette crise. C'est dans cet esprit, je le crois, que nous pouvons tous nous mobiliser.

par le DLA, qui les aide à bien répondre aux appels à projets. J'ai bien mesuré aussi, pour être précise, que les appels à projets, les AAP, sont moins faciles pour les acteurs de l'ESS que les appels à manifestation d'intérêt, les AMI. C'est aussi pour cela que j'ai souhaité très vite augmenter le DLA

je proposerai au Gouvernement que nous les prenions. Je le répète, ce rapport sera rendu fin avril, et j'aurai grand plaisir à le partager avec les sénateurs. L'IGF et l'IGAS sont mobilisées, et j'ai bien l'intention de consolider le modèle de la loi 2014, auquel je crois.

Conjuguant l'objectif de rentabilité, l'utilité sociale et le respect de l'environnement, l'ESS est devenue une référence en matière de développement économique durable. Le poids qu'elle représente dans l'économie globale ne cesse de s'accroître d'année en année. Mon département, les Hautes-Alpes, Mon département, les Hautes-Alpes, en offre une excellente illustration. C'est un territoire rural, où la proximité, la solidarité et la production locale de biens et de services reposent sur un grand nombre d'organisations coopératives, mutualistes et associatives, mobilisant à la fois des salariés et des bénévoles.

structure permettrait de soutenir directement les différents acteurs de l'ESS, tout en mettant en valeur leurs vertus sociales et écologiques dans l'économie concurrentielle. Par ailleurs, vous avez

l'économie sociale et solidaire fonctionne selon des règles de gestion souvent singulières, avec un engagement fort de celles et ceux qui en sont les animateurs. Parallèlement, elle souffre d'une grande difficulté à obtenir des financements à la mesure de ses besoins. C'est ce qui ressort des entretiens que j'ai eus avec de nombreux professionnels de l'ESS. Certes, des formules spécifiques de financement existent ; je pense notamment aux titres associatifs. Des formules ouvertes à d'autres secteurs économiques sont également susceptibles d'être utilisées, notamment les titres obligataires. Je n'ignore pas non plus que le secteur bancaire dispose de fonds ciblés pour le secteur de l'ESS.

comment pensez-vous contribuer concrètement à faire en sorte que, dans les territoires, les interlocuteurs des associations maîtrisent les outils de financement existants et puissent proposer une expertise technique pour les mettre en oeuvre et accompagner les acteurs de l'ESS dans leur financement ? prendre en compte, à terme, les spécificités de ce secteur et de ses besoins de financement par les investisseurs et l'ensemble du secteur bancaire ? À l'heure où l'épargne forcée des ménages serait devenue surabondante en raison de la crise du covid-19, ne serait-il pas envisageable d'orienter une partie de cette épargne vers l'ESS, qui participe à l'amélioration du bien-être et de la cohésion de notre société ? La parole est à Mme la secrétaire

ma question concerne l'inclusion des personnes en situation de handicap et leur orientation vers des entreprises adaptées, ou EA. Le Gouvernement a projeté de doubler, sur le quinquennat, le nombre de places en EA. Il a accéléré, en mai dernier, le déploiement de la plateforme « Mon Parcours Handicap », pour simplifier l'accès des personnes handicapées aux services adaptés. Ces initiatives vont dans le bon sens, mais il reste beaucoup de travail pour améliorer la fluidité des parcours.

de vous apporter une réponse. Pour ce qui est de vos deux premières questions, je veux rappeler, sur ce sujet qui me tient particulièrement à coeur, que le Gouvernement s'est engagé dans une politique volontariste et surtout pragmatique d'amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap, mais aussi de leurs proches.

une aide à l'embauche visant à favoriser l'emploi de ces personnes. Cette aide, d'un montant maximum de 4 000 euros, est attribuée aux entreprises et aux associations, quelles que soient leur taille et leur structure, qui auront embauché entre le 1 septembre 2020 et le 30 juin 2021 un salarié travailleur handicapé en CDI ou en CDD d'au moins trois mois rémunéré jusqu'à deux fois le SMIC. Parmi les mesures fléchées vers les entreprises adaptées, rappelons que 300 millions d'euros ont été déployés depuis l'été dernier, en direction de près de 5 000 entreprises sociales inclusives et, en particulier, de 800 entreprises adaptées. Ce plan a reçu 20 millions d'euros supplémentaires en décembre dernier, compte tenu du succès rencontré par ces projets créateurs d'emplois. Ce sont donc à ce

cela a déjà été rappelé, l'ESS représente un gisement colossal d'emplois durables, qui doivent participer à la relance économique, sociale, industrielle et écologique de notre pays. L'ESS démontre chaque jour que nous pouvons faire autrement, en plaçant l'humain au coeur de l'économie. En nous appuyant sur ce formidable réseau de compétences, d'action et de démocratie, nous pourrons apporter des solutions pertinentes à la crise sanitaire, écologique et économique.

Vous avez déjà évoqué les têtes de réseaux, qui ont pour mission d'accueillir, d'informer et d'accompagner. J'insiste sur la notion d'accompagnement et d'appui des structures, notamment en matière de levée de fonds et de développement commercial, compétences parfois peu représentées dans les organisations de l'ESS, ce qui tend à favoriser les plus grosses structures au détriment des plus petites. Cela s'est ressenti lors de la première séquence de la crise. Le Mouvement associatif a pointé la faible consommation par les associations des dispositifs mis à leur disposition pour les soutenir. pourquoi ne pas imaginer le développement d'un centre de formalité des entreprises dédié aux entreprises de l'ESS et géré par les Cress, à l'image de ce que font déjà les

2,5 millions de salariés travaillent dans ce secteur, soit 14 % des emplois en France. Avec la crise, et malgré une activité soutenue au premier trimestre de 2020, une nette chute a suivi. Entre juin 2019 et juin 2020, 52 500 emplois dans des coopératives, des mutuelles, des associations et des entreprises

Cette évolution inquiétante est majoritairement due au secteur associatif, qui perd plus de 7 % de ses établissements. Trois secteurs ont été particulièrement affectés : l'art et le spectacle, l'hébergement et la restauration, ainsi que le sport.

L'aide déployée par le mouvement associatif France Active doit permettre aux structures relevant de l'économie sociale et solidaire de poursuivre leur activité pendant la crise, de financer les emplois de leurs salariés et de pallier les difficultés liées à la trésorerie.

M. Michel Canevet. Madame la secrétaire d'État, la Bretagne est une terre particulièrement favorable à l'économie sociale, solidaire et responsable, notamment parce que l'on y trouve implantées beaucoup de coopératives, mais aussi de nombreux établissements mutualistes, des fondations et, bien sûr, nombre d'associations qui oeuvrent au quotidien pour aider au développement de la région et apporter un certain nombre de services à la population.

en matière d'éducation et de formation des jeunes. On sait qu'un certain nombre de ces derniers restent en difficulté, en marge du système éducatif traditionnel. Il importe de pouvoir leur apporter des réponses ; or il me semble que ce secteur d'activité est plutôt

j'ai demandé à la Banque de France, qui est mobilisée sur l'ESS, je vous l'ai dit, en lien avec les banques, de conduire des travaux statistiques pour suivre les évolutions de l'arrêté de 2020, qui prévoit que la quote-part minimale égale à 5 % de l'épargne non réglementée soit allouée à l'ESS. Nous étudierons l'intérêt de porter ce seuil de 5 % à 10

Loire, près de 800 emplois ont été détruits en Maine-et-Loire et 3 500 dans l'ensemble de la région en un an. L'ESS est un secteur qui reste fragile. Nous avons évoqué l'ESS à l'échelon national, mais c'est également un sujet européen. L'ESS représente en effet près de 20 millions d'emplois dans l'Union européenne et environ 9 % de la population active du continent. Les 26 et 27 mai 2021 aura lieu le Sommet européen de l'économie sociale

qui ne défendent pas les valeurs des acteurs de l'ESS : la démocratie, la lutte contre les inégalités sociales, l'intérêt général et la transformation économique et écologique. Lors d'une interview au journal en novembre 2020,

va prendre la présidence de l'Union européenne en 2022 et se doit d'être au rendez-vous et à la hauteur des enjeux. La

Ce plan d'action est en cours d'écriture- un point d'étape sera réalisé à Mannheim au mois de mai -, et il prendra forme définitivement à l'entrée de l'hiver, en octobre ou en novembre 2021.

madame la secrétaire d'État, de ces réponses. L'ESS représente un véritable espoir. Nos territoires le savent bien. L'ESS peut incarner le monde d'après et l'économie de demain. Il faut que ce modèle soit étendu à l'échelon européen. On espère que la France sera à la hauteur des enjeux.

l'ESS peut être au coeur de la transformation de notre économie : elle peut favoriser les transitions vers des modèles plus résilients en matière écologique, économique et sociale, en s'appuyant sur leur potentiel démocratique et de coopération. coopération. Il faut soutenir les entreprises de l'ESS en faveur de la transition sociale et écologique. Il faut soutenir le développement de l'ESS dans un contexte marqué par la crise sanitaire, économique et sociale et formuler des propositions en ce sens. Cela va sans dire,

L'implantation de l'ESS dans le secteur des déchets et de l'économie circulaire a permis ces dernières années d'accélérer les transitions en matière de consommation. Dans la seule filière textile, les tonnages de déchets collectés ont été multipliés par trois ans et sont passés de 75 000 tonnes en 2008 à 250 000 tonnes en 2019. L'ESS occupe une place importante dans cette filière puisqu'elle gère 36 centres de tri sur les 63 existants. Je pense par exemple aux activités du Relais et d'Emmaüs, etc. Le réseau Envie, quant à lui, qui compte une soixantaine d'établissements en France, collecte entre 25 % et 30 % des déchets d'équipements électriques et électroniques en France et rénove plus de 120 000 appareils par an.

Transversales par définition, les difficultés en matière d'accès au logement ont des conséquences directes dans les domaines de l'éducation, de l'intégration et de l'insertion professionnelle.

Cette triste réalité nous rappelle que, si ce sujet est régulièrement évoqué et pris en compte par les décideurs publics, nous n'avons pas encore trouvé de baguette magique afin d'enrayer ce triste constat. En 2007, l'association Toit à moi a été créée, afin de venir en aide aux personnes sans domicile fixe. Partant du constat qu'une association est bien plus efficiente si elle est propriétaire des logements qu'elle propose aux plus démunis, mis en oeuvre un principe simple pour lever des fonds, certes modestes, mais tout de même : si cent personnes donnent 20 euros par mois pendant cinq ans, l'association devient propriétaire d'un logement à l'issue de cette période, les donateurs pouvant bénéficier d'une réduction fiscale. Ainsi, cette association s'est constituée au fil des années un parc immobilier, certes modeste comparé à celui d'un bailleur social, mais qui lui permet de répondre, à son échelle, à la demande de logement des sans-abri d'un

Marta de Cidrac. Madame la secrétaire d'État, l'insertion professionnelle des jeunes est l'un des piliers fondateurs de l'économie sociale et solidaire. Cette importance a été reconnue dans le cadre du plan de relance puisque la moitié des sommes engagées pour le secteur sont dédiées à l'insertion. est important, mais nécessaire, quand on sait combien l'ESS est une manière concrète de faire vivre l'égalité des chances. Cette branche permet en effet aux jeunes de faire leurs preuves dans un cadre adapté. Dans le seul département des Yvelines, on dénombre plus de 40 structures d'insertion par l'activité économique, représentant 900 salariés. Bien d'autres structures de l'ESS mettent en oeuvre des démarches de lutte contre l'exclusion. Cependant, elles se révèlent bien souvent fragiles du fait de leur modèle économique. La question de leur pérennité économique se pose pour la grande majorité des projets, à juste titre, car peu de structures tendent malheureusement vers cet horizon. Si les entreprises et les associations de l'ESS reconnaissent l'effort fait par le Gouvernement, elles pointent aussi un manque de cohérence globale et quelques trous dans la raquette. Deux points sont régulièrement mentionnés d'une part, le besoin d'attirer les jeunes plus qualifiés afin de bénéficier de leurs compétences ; d'autre part, les difficultés de trésorerie au-delà de la période de crise actuelle, pour lesquelles il faut trouver des solutions pérennes. Il convient donc de répondre aux difficultés structurelles de l'ESS tout en poursuivant la dynamique pour l'insertion des jeunes, des plus éloignés de l'emploi. Madame la secrétaire d'État, comment comptez-vous accentuer le lien entre les structures de l'ASS et les services de l'emploi-

Les missions locales qui oeuvrent pour l'accompagnement de nos jeunes aujourd'hui bénéficient de 190 millions d'euros au sein du plan de relance.

Actuellement, l'Éducation nationale semble faire de l'ESS davantage un objet de découverte qu'un élément de programme. Ainsi, du 22 au 27 mars prochain sera organisée en France la semaine de l'économie et solidaire à l'école. Différentes ressources seront mises à la disposition des enseignants et des lycéens, comme un dossier pédagogique et des fiches pratiques. Cette présentation de l'ESS s'inscrit plus dans une logique d'initiation que dans une logique d'enseignement, au travers du parcours d'avenir, qui permet aux élèves, de la sixième à la terminale, de construire progressivement, et tout au long de leurs études secondaires, une véritable compétence à s'orienter. À un moment où la préoccupation majeure de la France est l'accès de ces jeunes au travail, ne serait-il pas préférable d'inscrire l'économie sociale et solidaire dans le programme des élèves de la seconde à la terminale, pour en faire un enseignement de base, de nature à renforcer leur insertion dans la vie professionnelle et à susciter des vocations ? J'ai

Comme vous le savez, un certain nombre de ces structures de l'économie sociale et solidaire intervenant dans le secteur du réemploi et de la réutilisation connaissent ou vont connaître des difficultés financières importantes. Elles disposent bien souvent d'une trésorerie insuffisante ou de fonds propres trop faibles pour affronter les conséquences de la pandémie de la covid-19.

a prévu la mise en place de nouveaux fonds par les éco-organismes à des filières à responsabilité élargie des producteurs. Les filières qui produisent des produits électriques ou électroniques, des meubles ou des articles de bricolage ou de jardinage devront y participer à hauteur de 5 % de leur écocontribution. devrait représenter une enveloppe de 30 millions d'euros à destination des recycleries, ressourceries et autres structures de l'ESS. Le décret du 27 novembre 2020 qui met en oeuvre ces dispositions de la loi AGEC prévoit une attribution des financements sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible

de proximité : la fixation d'une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit et celui de la réalisation des opérations garantissant que ces aides bénéficient aux petites entreprises locales, même hors ESS. J'entends la crainte des différents acteurs associatifs,

Je poursuis actuellement les discussions avec le ministère de la transition écologique pour définir comment nous assurer au mieux du fléchage nécessaire. S'il faut

Comment faire de l'ESS un levier majeur, peut-être la clé de voûte de la relance économique, en tout cas d'une certaine relance économique, celle du « monde d'après », dans une logique de résilience, d'innovation et de coopération

Il est nécessaire que ces valeurs fondamentales demeurent présentes et actives au sein de toutes les entreprises de l'ESS. Le principe de la lucrativité limitée, c'est-à-dire la mise au service des hommes et du développement de projets des excédents, donc des bénéfices dégagés, la rémunération limitée ou nulle du capital

soulignent l'importance de s'inspirer des principes et pratiques de l'ESS pour reconstruire un monde durable, afin de créer ce nouveau paradigme économique appuyé sur les logiques de l'économie circulaire, de la sécurité alimentaire, de l'échange de bonnes pratiques, du développement économique local, de l'innovation sociale et du bien commun. L'ESS, c'est vert, c'est durable et c'est humain ! La plupart des entreprises de l'ESS s'appuient sur leurs membres, sont ancrées dans leur communauté, où elles jouent un rôle essentiel dans le développement économique et la gouvernance locale. Ainsi, dans le cadre de la relance, l'ESS peut favoriser la création d'emplois décents, mais aussi un développement plus centré sur les personnes à l'échelon local. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire visent plutôt à fournir des biens et des services à leurs membres et aux communautés dont elles sont proches. Elles sont souvent dirigées ou détenues par ces communautés, donc enclines à relever à la fois les défis du changement climatique et de la réduction de la pauvreté. Le Gouvernement devrait inclure les ESS dans la conception et la mise en oeuvre des mesures d'intervention et de reconstruction. Il est nécessaire de saisir les occasions de passer à des économies plurielles qui incluent et promeuvent des modèles d'entreprises alternatifs orientés vers la personne et la planète. Les politiques publiques visant à créer et renforcer des écosystèmes pour l'ESS sont décisives pour pouvoir mettre en place un programme de développement transformateur de notre modèle économique et social, donc de notre société.